Les articles 44 et 49 du projet de loi PACTE sont les deux articles clés permettant la privatisation d'ADP. Par cohérence avec leur suppression, il serait souhaitable de supprimer également les articles 45, 46 et 50.

Ainsi modifiés, ces articles conserveraient leur pertinence, même si ADP restait publique, et pourraient servir de base de travail utile aux députés en nouvelle lecture si ces derniers veulent améliorer la régulation économique de l'entreprise avant de la privatiser. Je ne comprends

Madame la présidente, autant je respecte la présidence de la commission spéciale, autant il revient au service de la séance de nous dire quels amendements et articles « tombent

de voter la suppression

Au vu de ce qui s'est passé avec les recettes de la taxe carbone, dont tout le monde savait qu'elles seraient affectées non pas à la transition énergétique, mais au budget de l'État, on peut se demander si cette cession d'actifs ne subira pas le même sort. Pour vous citer encore une fois, toujours le 8 mars 2018, vous avez déclaré : « Ce n'est pas le rôle de l'État que de recueillir régulièrement des dividendes au lieu d'investir dans l'avenir des Français. » Alors, je vous prends au mot, monsieur le ministre : l'État n'a peut-être pas pour vocation à recevoir des dividendes, mais il doit rester un actionnaire stratégique pour nos territoires. territoires. Précisément, les investissements pour l'avenir des Français que vous avez évoqués ne pourraient-ils pas être financés par ces mêmes dividendes, afin de maintenir des services publics gratuits en milieu rural, par exemple ? Ce maintien est d'ailleurs l'une des multiples revendications exprimées par nos concitoyens à l'occasion du grand débat national. Pour l'heure, votre gestion de ce dossier est préjudiciable à notre économie et à l'avenir des Français. Si vous décidez de ne pas revenir sur la privatisation d'ADP, comme vous en avez l'intention, vous devrez assumer la responsabilité de votre vision à court terme de l'État stratège. La seule question que nous devons nous poser est la suivante : l'État stratège que vous prétendez représenter assure-t-il une bonne gestion avec un tel projet ? Cet enjeu mérite un autre débat que celui qui est lié à un article noyé dans le présent projet de loi ! La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann,

... À partir du moment où le Sénat a décidé d'annuler cette privatisation, je ne vois pas pourquoi nous passerions beaucoup de temps à réfléchir sur la régulation d'un processus dont il ne veut pas et dont l'examen reviendra à l'Assemblée nationale.

Lienemann, pour explication de vote.

Le débat politique est intéressant, dans la mesure où chacun prend ses responsabilités ! Les sénateurs ont pris les leurs et ont choisi, dans une curieuse alliance entre le parti socialiste, le parti communiste et Les Républicains, de s'opposer

pas cohérent ! Comme le disait très bien le sénateur Bourquin, le surréalisme a ses limites. Nous sommes au Sénat, pas dans un atelier de surréalisme ! Et je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange à vouloir discuter des conséquences d'une décision que vous n'avez pas voulu prendre.

Fabien Gay, pour explication de vote.

propose de consacrer 20 % des bénéfices liés aux activités commerciales au financement de ces infrastructures. C'est un progrès par rapport à la situation

Pour la démocratie, madame la sénatrice, il n'est pas bon non plus d'accuser un ministre de chantage, et tel n'était pas du tout mon propos. Et vous le savez parfaitement.

: « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. » C'est votre seule option, monsieur le ministre.

et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

aéronautique. La privatisation de la gestion des aérodromes a entraîné une hausse des redevances aéroportuaires et a provoqué la disparition de certaines de ces structures. Il est donc proposé de préciser

critère d'intérêt général reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, étant précisé qu'il doit y avoir rattachement à une association reconnue d'utilité publique et affiliation des aéroclubs à la Fédération française aéronautique.

pour ADP, quelle que soit la décision finale du Gouvernement.

attendent un régulateur indépendant qui soit capable de donner son avis sur la juste rémunération des capitaux investis, lors de l'homologation annuelle des tarifs. C'est un pas en

Quel est l'avis de la commission

puisqu'il vise à rétablir l'autorisation de transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux. Après avoir passé un peu de temps sur Aéroports de Paris et sur l'encadrement d'une l'encadrement d'une privatisation dont le Sénat ne veut pas, nous allons maintenant avoir une discussion sur le rétablissement d'une privatisation dont le Sénat voudra

Monier, pour explication de vote. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux attirer votre attention sur une autre problématique que poserait la privatisation de cette entreprise publique

que vaut un ticket à gratter, 1,04 revenait à l'État et 1,5 était destiné à la Fondation du patrimoine. Après la privatisation, de telles opérations seront-elles encore possibles ? Aucune garantie n'est apportée quant à la répartition des sommes qui seront affectées au secteur patrimonial lors de futures éditions. La FDJ participe au financement de plusieurs secteurs, notamment, mon collègue, celui du sport, mais aussi celui du patrimoine des taxes affectées provenant des mises des joueurs. Cette implication singulière est particulièrement importante. Monsieur le ministre, comment comptez-vous garantir que le nouvel investisseur privé accordera au patrimoine et au sport une attention aussi forte que la Française des jeux, contrôlée par l'État ? Si l'État n'est plus majoritaire, il n'y aura plus les mêmes marges de manoeuvre ni des moyens de pression comparables pour défendre les secteurs que la FDJ finance actuellement et pour lesquels, on le sait, les pouvoirs publics se désengagent de plus en plus, faute de budget suffisant. Il convient donc de ne pas remettre en cause les différentes ressources financières affectées au patrimoine et de ne pas porter un mauvais coup à la nécessaire régulation républicaine des jeux d'argent. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

En effet, la Française des jeux prend appui sur un réseau de plus de 30 000 points de vente, qui sont des bars, des tabacs, des magasins de journaux. Répartis sur plus de 11 000 communes, pour bon nombre d'entre eux, le dernier commerce en milieu rural. La Française des jeux mobilise annuellement plus de 780 millions d'euros pour rétribuer les détaillants, ce qui représente un complément de chiffre d'affaires de plus de 25 000 euros par point de vente et par an, une somme qui contribue largement à la viabilité de ces petits commerces. Les relations entre la Française des jeux et ses détaillants reposent sur une base contractuelle qui permet une rétribution à hauteur d'un taux d'environ 5,5 sur le chiffre d'affaires des jeux. Ces relations sont à la fois bonnes et fragiles, car la stratégie repose sur des points de vente physiques et sur une forte implication des revendeurs. Qu'en serait-il demain ? La future gouvernance n'aurait-elle pas, pour maximiser ses bénéfices, tendance à durcir ses relations avec les buralistes ? Le développement des nouvelles technologies ne va-t-il pas favoriser le recours à des jeux dématérialisés qui sont très lucratifs ? Face à ces interrogations, le maintien de la gouvernance de la Française des jeux dans le giron public me semble être une garantie en termes d'aménagement du territoire pour continuer à conforter la présence de ces points de vente, notamment en milieu rural. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Je suis satisfait que la commission spéciale ait choisi de s'opposer à cette privatisation et je partage les réserves de ceux qui se sont exprimés dans le

s'élèveraient à 62 % du produit brut des jeux, alors que l'État prélevait auparavant 9,3 % des mises. Ce n'est pas du tout un jeu à somme nulle ! Beaucoup craignent d'ailleurs que des opérateurs aujourd'hui rentables ne fassent faillite.

Nous ne devons cependant pas oublier que le jeu n'est pas une marchandise comme les autres. Je veux revenir à mon tour sur la question des addictions. L'Observatoire des jeux et de nombreuses associations qui oeuvrent avec beaucoup de pugnacité contre les addictions nous alertent sur l'évolution du nombre de joueurs à risque excessif- 300 000 -et sur l'augmentation assez forte du nombre de joueurs à risque modéré. Ces joueurs ne compromettent pas l'équilibre de leur budget quotidien en jouant de façon pathologique, excessive, mais leur nombre augmente et atteindrait aujourd'hui 1 million dans notre pays, ce qui doit nous conduire

obtenir de l'argent en privatisant, mais je crains que nous n'en dépensions bien davantage pour essayer de lutter contre les addictions. Il faut donc une politique publique de jeu responsable.

l'accès au privé de manière à libérer les capacités à s'ouvrir au monde extérieur et à accélérer sa montée en compétences. Quand on connaît les réalités du monde extérieur en matière de jeux, c'est un peu inquiétant

nier totalement la loi de 2010, qui soulignait les risques d'une déstabilisation économique des filières concernées, dont mon collègue Vogel a parlé, notamment les paris hippiques et le PMU. Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, nous avons des motifs d'être inquiets inquiets quant à l'avenir des jeux, des filières et des emplois sur l'ensemble de nos territoires.

En revanche, qu'il y ait un vrai sujet sur la régulation, le contrôle des jeux et l'addiction au jeu, j'en suis parfaitement d'accord et je partage tout ce qui a été dit sur l'ensemble des travées du Sénat. Oui, il faut lutter contre l'addiction au jeu

Il a intérêt à la fois à commercialiser au maximum les jeux et à rendre les Français les plus addictifs possible aux jeux qu'il commercialise puisqu'il est acteur de cette commercialisation et que cela garantit la rentabilité de son activité ! Et puis, de l'autre côté, il se décale et il essaie de réguler et de contrôler le plus possible. Là encore, je pense que le Gouvernement a une position cohérente : si on veut lutter contre l'addiction au jeu, il ne faut pas que l'État soit juge et partie en la matière. Il faut qu'il régule, il ne faut pas qu'il commercialise. Je vous invite à réfléchir à cet argument. Je pense que tous ceux qui, dans cette enceinte, sont attachés à l'État régulateur, comme je le suis, estimeront qu'il ne peut pas être celui qui commercialise et celui qui régule.

Il est évident que ce qui compte dans la Française des jeux, ce ne sont pas les dividendes, lesquelles sont inférieurs à 100 millions d'euros, mais les revenus de la fiscalité qui sont supérieurs à 3 milliards d'euros. Comme ministre des finances, entre 100 millions d'euros et 3 milliards d'euros, j'ai toujours préféré les 3 milliards ! C'est

jeux. L'opération que nous vous proposons consiste à permettre à l'État de conserver 20 % dans le chiffre d'affaires de la société. Il serait actionnaire à hauteur d'environ 20 %, de façon à pouvoir pérenniser les dividendes de ces associations d'anciens combattants. C'est un engagement que nous prenons, qui est garanti par le maintien de la présence de l'État au conseil d'administration de la société. S'agissant des buralistes, nous faisons évidemment très

Nous garantirons par la convention qui sera signée entre l'État et la future société d'exploitation de la Française des jeux la pérennisation des activités du loto du patrimoine. C'est un engagement que je prends devant vous et que je prendrai envers Stéphane Bern. Le loto du patrimoine est un succès auquel Stéphane Bern a contribué. Nous devons garantir noir sur blanc dans cette convention le maintien du loto du patrimoine.

car personne n'a envie de voir se développer l'addiction au jeu, en particulier chez les jeunes, en France. Je suis tout aussi sensible que vous à ce sujet. Vous me permettrez d'observer que la situation actuelle n'est pas satisfaisante,

D'abord, elle reviendra à une autorité administrative indépendante de régulation et de surveillance des jeux d'argent et de hasard qui sera dotée d'une compétence générale sur les jeux en ligne, les jeux sous droits exclusifs de la Française des jeux et du PMU. Cette autorité administrative indépendante aura vocation à contrôler les points de vente en second niveau. Ce sont les opérateurs qui contrôleront en premier niveau, mais au second niveau, cette autorité sera chargée de vérifier l'effectivité et la rigueur des contrôles assurés par les opérateurs. Elle disposera à cette fin de tous les rapports, de tous les résultats des inspections des points de vente. Elle devra informer les ministères compétents en cas d'abus ou de manquement des détaillants.

par arrêté. Ce point est capital. Ce n'est pas le futur opérateur privé qui va déterminer les taux de retour aux joueurs qui définissent l'addiction. Il reviendra à un arrêté de définir ces taux de retour aux joueurs qui seront ensuite affectés jeu par jeu.

que l'autorité administrative de contrôle déterminera les jeux autorisés dans la gamme définie par l'État en fonction du taux de retour aux joueurs déterminé par arrêté. est conditionnalité de l'addiction, c'est-à-dire le taux de retour et le type de jeu, reste du domaine et de la compétence du secteur public. Tout ce qui est contrôle de cette régulation, bon fonctionnement des opérateurs et respect des règles relève du contrôle de cette autorité

observations. D'abord, l'alibi de la simplification et de l'alignement sert souvent à justifier la dérégulation d'un certain nombre d'institutions.

Elle sécurisera le niveau et la dynamique des prélèvements publics sans accroître la pression fiscale sur la Française des jeux. Nous avons donc découpé l'activité de cette dernière en quatre segments distincts : les paris sportifs en ligne, les paris sportifs en points de vente, les jeux de tirage traditionnels et les autres jeux de loterie.

L'activité de paris sportifs présente une spécificité en ce qu'elle est exercée par la Française des jeux sous monopole pour les paris en points de vente, mais de façon concurrentielle pour les paris sportifs en ligne.

deuxièmement, d'ajuster le taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne et, troisièmement, d'ajuster le taux de prélèvement sur les paris sportifs en réseau physique de distribution.

rejeté la privatisation, mais cela ne nous empêche pas de travailler sur la fiscalité, preuve de la bonne volonté, du sérieux et du travail de notre assemblée.

D'abord, cette réforme ne préjuge pas l'avenir de la Française des jeux. Il s'agit d'une actualisation bienvenue d'un régime fiscal obsolète. Ensuite, le changement d'assiette se traduira par un rendement équivalent et un dynamisme préservé des recettes. Les recettes destinées à soutenir le mouvement sportif sont sécurisées

: sa restauration génère une économie touristique qui, dans les territoires ruraux, permet de maintenir une activité commerciale et des activités de service. Je suis présidente d'une association qui regroupe 160 petites cités de caractère de France.

Martial Bourquin, pour explication de vote.

du Gouvernement et des collectivités pour y parvenir, mais on a aussi besoin du loto du patrimoine.

français -, mais si on laissait tomber tout ce patrimoine extraordinaire, cette mosaïque formidable de vieilles pierres de nos territoires, on ferait une erreur colossale

Ce n'est pas parce qu'on essaie de défendre les comptes de la Nation qu'on n'est pas attaché au patrimoine. Je considère que le loto du patrimoine est un vrai succès. Je répète à M. Bourquin, qui s'en inquiétait,

partageons le souci du Gouvernement de protéger les mineurs face aux jeux d'argent et de hasard. Toutefois, la disposition proposée n'a pas de lien avec le présent projet de loi, qui porte sur la croissance et la transformation des entreprises.

Je vous remercie